J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la fin de 2020, la France devrait avoir construit 100 000 logements de moins qu'en 2019, soit une réduction d'environ 25 % de la production annuelle. Après la crise sanitaire, dont nous ne sommes peut-être pas sortis, c'est une crise aiguë du logement qui s'annonce. Ce chiffre, avancé par la Fédération des promoteurs immobiliers de France et certains observateurs, s'explique par l'arrêt du secteur de la construction pendant presque un trimestre. cette prévision ne se réalisera pas, monsieur le ministre, mais elle souligne en tout cas la gravité de la situation et l'urgence d'y apporter des remèdes appropriés. Si nous sommes bien dans l'urgence, prenons pourtant le temps de porter le bon diagnostic sur la maladie. Le secteur immobilier s'inscrit dans le temps long, les logements neufs et réhabilités ne représentant, chaque année, guère plus de 2 % des logements existants. Plus que dans d'autres domaines, les décisions d'aujourd'hui auront un impact sur les décennies à venir. Il nous faut donc tirer les bonnes leçons de la crise. Le logement y est apparu comme un bien de première nécessité. Sans toit pour sa famille, il est impossible de se protéger de l'adversité et de se projeter dans l'avenir. À cet égard, le confinement a mis en évidence une grande inégalité entre les Français. Selon une récente étude de l'Insee, 5 millions de personnes vivent dans un logement suroccupé. Nos concitoyens ont d'autant plus mal vécu cette épreuve qu'ils sont mal logés. Or cette situation va s'aggraver dans les prochains mois, nous mettant au défi de rattraper le temps perdu et de construire plus. La crise du logement sera d'autant plus dure que la crise sanitaire a laissé la place à une crise sociale et économique. La Banque de France a indiqué qu'il y aurait vraisemblablement plus d'un million de chômeurs de plus début 2021 qu'il y en avait fin 2019. Cela va se traduire

Par ailleurs, en raison du développement massif du télétravail, le marché de l'immobilier professionnel pourrait connaître un tournant, ouvrant la voie à une reconversion de nombreux bureaux en logements. De même, les investisseurs institutionnels pourraient revenir sur le marché du logement résidentiel. C'est une opportunité qu'il nous faut en tout cas saisir. Construire plus, plus abordable, mais aussi construire mieux et plus durable. En effet, la crise sanitaire ne doit pas masquer les enjeux climatiques et environnementaux, qui rendent impérieuses la rénovation thermique des bâtiments et une réelle sobriété foncière. Construire mieux, c'est également prendre en compte que, à l'instar du choléra et de la tuberculose, qui ont façonné la ville haussmannienne du XIXsiècle, le Covid-19 va modifier la ville de demain. Compte tenu de l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est moins une « ville jardin » qu'une ville compacte qualitative, où proximité rime avec solidarité et espaces partagés, Enfin, il ne sera pas possible d'atteindre ces objectifs sans tenir compte d'un tissu économique durement éprouvé par la crise. Beaucoup d'entreprises sont menacées de faillite ; or, dans la chaîne du logement, chaque maillon est solidaire. Pour qu'il n'y ait pas de rupture aujourd'hui, il nous faut mettre en oeuvre une chaîne de loyauté économique, pour prendre en charge les surcoûts et les retards. Pour que cette chaîne soit plus résiliente demain, nous devrons faire confiance aux acteurs économiques et libérer les énergies.

qu'il faut nous appuyer sur trois acteurs : les bailleurs sociaux, Action Logement et les investisseurs institutionnels. Les bailleurs sociaux sont prêts à jouer leur rôle de filets de sécurité, mais nous devons pour cela leur redonner les moyens d'agir, de construire,

une TVA à 5,5 %, c'est 5 000 euros de moins par logement, ce qui est déterminant quand on parle de 130 000 constructions neuves et de 150 000 rénovations par an. Action Logement, ensuite, doit être replacée au centre du dispositif. Le groupe paritaire est actuellement contesté dans son existence, dans ses objectifs, et il doit se recentrer sur sa mission première, qui est de loger les salariés, car ils en ont absolument besoin. besoin. Enfin, il faut faire revenir les investisseurs institutionnels dans le logement. C'est sans doute là que doit porter l'effort pour réussir à construire plusieurs dizaines de milliers de logements en plus chaque année. Pour les accompagner, il est nécessaire de faciliter la conversion des bureaux en logements, soit en jouant sur les délais, soit en sécurisant le taux réduit de TVA. Il est également impératif de considérer l'investissement dans le logement comme un investissement productif économiquement et socialement. J'ai la conviction qu'il faut libérer les énergies. Fixons-nous l'objectif d'une division par deux des délais des procédures et des recours, car le logement souffre de la complexité excessive du droit de l'urbanisme. Il faut aujourd'hui

C'est pourquoi je vous propose, monsieur le ministre, de réunir autour de vous, dès cet été, un « Ségur de la simplification du droit de l'urbanisme » pour aboutir à des propositions partagées et juridiquement sûres, qui permettront de réussir durablement la relance de la construction.

Soyons pragmatiques : en cette période de crise économique et de chômage, incitons ceux qui en ont les moyens à vider leur « bas de laine » pour leur logement. Monsieur le ministre, proposez

Le troisième défi sera de préserver l'accès et le maintien dans le logement. Le maintien dans le logement, c'est la prévention des impayés. Encore une fois, je veux vous alerter, monsieur le ministre, sur la grande disparité des situations selon les départements et les métropoles. L'État doit se réinvestir dans le Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Je crois que la proposition de la Fondation Abbé Pierre d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour l'aide à la quittance doit en tout cas être étudiée pour pouvoir agir dès que nécessaire. Accéder au logement, c'est aussi maintenir la possibilité d'une accession sociale, malgré la crise et malgré la hausse des prix du foncier. L'APL accession et le prêt à taux zéro (PTZ) sont des outils qui manquent, même s'il faut les adapter aux exigences de sobriété foncière. Enfin, nous devons aussi développer deux autres dispositifs deux autres dispositifs qui ont fait leurs preuves, à savoir les organismes de foncier solidaire et les « chartes promoteurs », en les sécurisant et en les élargissant. Monsieur le ministre, j'espère que ces quelques propositions permettront de faire prendre un nouveau départ au secteur du logement et du bâtiment.

Avant de revenir sur la situation actuelle et de répondre aux différentes questions que vous avez abordées, permettez-moi tout d'abord de poser un diagnostic, qui est, je le sais, partagé sur les travées de cet hémicycle, sur les effets de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire a d'abord mis en exergue les nombreuses inégalités : inégalités sociales, inégalités territoriales. On les connaissait, mais elles ont été une fois de plus mises très fortement en évidence, certains ménages, qui en avaient la possibilité, quittant les métropoles pour aller dans leurs résidences secondaires, d'autres vivant le confinement dans des endroits beaucoup plus exigus et, parfois, dans le mal-logement. Le confinement et le télétravail ont aussi montré les difficultés de certains ménages face non seulement à la mauvaise qualité de leur logement, mais aussi, parfois, à leur mauvaise connexion. Le télétravail n'était pas une réalité pour tous nos concitoyens. Le facteur numérique, qui, nous l'avons souvent dit, était là pour résoudre les inégalités territoriales, bien souvent, trop souvent, et encore aujourd'hui, n'a fait que les accroître. Quelles sont les conséquences que nous devons tirer de cette période ? Je voudrais axer mon propos sur quatre principaux points, répondant ainsi à un certain nombre de vos questions. Le premier axe, c'est d'aller le plus loin possible sur la rénovation du bâtiment. Le rapport de la commission des affaires économiques met bien cet objectif en avant, soulignant que les Français sont inégaux face au logement ; dans cette inégalité, il y a la question de la rénovation des logements.

en activité depuis le 1 janvier, permet de répondre à un certain nombre de ces besoins. D'abord, parce qu'elle est très simple d'accès. Ensuite, parce que c'est une prime qui est sociale

Le deuxième axe, c'est de soutenir le secteur de la construction. La priorité du Gouvernement en ce moment, comme vous le savez, c'est la question de l'emploi. Or le secteur de la construction, c'est plus de 2 millions d'emplois. L'objectif est clair : il faut poursuivre la construction de logements abordables. avons besoin de deux choses. D'abord, et vous l'avez très justement dit, madame la sénatrice, il faut absolument soutenir les entreprises du bâtiment, sachant que le secteur du logement est un chaînon dont

la commande sur les territoires. Le fait d'abonder à hauteur de 1 milliard d'euros la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dans le prochain texte financier va dans ce sens, mais il nous faut aller plus loin. J'ai demandé, par exemple, à toutes les agences dont j'ai la responsabilité de mettre en oeuvre les projets d'ores et déjà décidés et de ne rien décaler. J'ai demandé également à l'ensemble de mes équipes d'être des facilitateurs. On sait, encore aujourd'hui, que ce qui relève de l'instruction des services de l'État met parfois trop de temps. Il faut donc être plus rapide. L'envie,

ou la lutte contre les logements vacants. Tels sont les trois axes,, que j'ai fixés comme priorité d'action à mes équipes au lendemain de la crise sanitaire s'agissant des modifications de l'aménagement du territoire. Enfin, puisque que le temps m'est compté, j'aborde un quatrième objectif : la réponse à la crise doit être évidemment sanitaire, d'abord, économique, pour préserver les emplois, mais il s'agit aussi d'éviter une crise sociale. À ce titre, le logement a une part fondamentale dans tout ce que nous allons faire. Nous allons d'abord accompagner les ménages qui en ont besoin pour payer leurs loyers. On pourra reparler du FSL, mais j'attire votre attention sur la décision des partenaires sociaux de créer une aide spécifique d'Action Logement, avec qui j'ai plaisir à travailler tous les jours, d'un montant de 150 euros par mois pendant deux mois les familles qui voient leur reste à charge profondément augmenter, s'agissant de leur loyer, soit parce que leurs revenus ont diminué, soit parce que leurs dépenses ont augmenté. Il s'agit également d'accompagner la production de logements sociaux. Je n'entre pas dans le détail des mesures, qui portent sur la TVA ou d'autres aspects, mais nous aurons aussi ce débat lors des

en deux ans, 2018 et 2019, ce sont 150 000 personnes que nous avons sorties d'un logement très insalubre ou de la rue pour leur donner un vrai « chez-soi ». Il faut conclure, monsieur le ministre. Vous avez très largement dépassé votre temps je dirai que c'est évidemment avec grand plaisir que je travaillerai avec vous sur la simplification. N'oubliez pas que nous sommes même en en train de réécrire le code de la construction pour passer d'une simplification à une réforme totale, puisque nous ne mettrons que les objectifs, sans donner les chemins à parcourir. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour.

mais aussi sur les communes, leur capacité à accompagner cette production en la finançant, en accueillant les nouvelles populations. Je pense notamment aux communes qui sont soumises à l'article 55 de la loi du Les préfets de région auraient dû réunir au printemps les commissions appelées à statuer sur le sort des communes qui n'ont pas atteint leurs objectifs ; on sait que, la marche devenant de plus en plus haute, elles devraient être plus nombreuses. Ces commissions ne se sont finalement pas réunies, mais elles devraient le faire prochainement. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, si vous allez donner des instructions pour que les préfets de région prennent en compte les situations dans lesquelles ces communes vont se trouver avec la baisse de recettes qu'elles vont subir en 2020, et peut-être ultérieurement. Et puis, il y a la période triennale à venir, soit 2020, 2021 2022. Pour 2020, tout le monde l'a dit, on va avoir, si ce n'est une année blanche, en tout cas une année fortement impactée

de logements, qui seront dans des situations extrêmement compliquées. Monsieur le ministre, je ne vous parle pas des quelques communes qui « ont les moyens » de ne pas faire, parce qu'elles ne veulent pas faire ; je vous parle de toutes les autres. Nous savons tous ici que l'objectif de 2025 était déjà inatteignable pour beaucoup. Avec la nouvelle situation, cela va devenir mission impossible. Ne serait-il pas temps de remettre tout cela à plat et de voir comment, contractuellement, on pourrait accompagner toutes ces communes soumises à l'article 55 qui vont avoir beaucoup de difficultés à faire ce que la République leur demande de faire ?

mettre à plat l'évolution de leurs données financières. J'attire votre attention sur un dispositif dont on a beaucoup parlé ici, à savoir les titres participatifs, que Mme la sénatrice Estrosi Sassone a beaucoup défendus. Ils marchent incroyablement bien et ont été certainement

je vous confirme effectivement que je n'avais volontairement pas donné instruction aux préfets de réunir des exécutifs locaux avant que les élections municipales ne soient terminées. J'ai signé la circulaire voilà tout juste quelques jours pour fixer un calendrier un calendrier de réunion de ces commissions à partir du 30 juin. Effectivement, les délais vont être plus serrés que d'habitude, mais je pense que vous auriez fait la même chose à ma place : il n'était pas concevable de commencer à faire ses consultations avant les élections municipales. Évidemment, dans cet échange contradictoire, j'ai demandé

déjà beaucoup discuté ici ? Je me souviens notamment de l'illustre amendement Daubresse sur la question, qui a fait beaucoup débat, et qui a permis de faire une première évolution. Je pense également à ce que nous avions fait dans les communes d'Île-de-France.

Nous serons tous obligés de constater que nous n'avons pas pu faire. Cherchons plutôt à voir comment accompagner les communes et les bailleurs sociaux plutôt que de les mettre dans un, parce que cela va décourager certains, qui avaient peut-être envie de faire et qui se diront : « Après tout, ce n'est plus la peine

pour leur permettre de conserver leur logement, tant dans le parc privé que dans le parc public, d'ailleurs. Dominique Estrosi Sassone vient d'exposer les grandes lignes de notre rapport commun à la commission des affaires économiques, et je l'en remercie vivement. Monsieur le ministre, il faut également réinterroger les politiques publiques à l'oeuvre, comme sur l'hébergement et les structures collectives, la rénovation énergétique, l'ambition d'une politique de société pour la politique de la ville, l'augmentation de la production de l'offre. Si le logement est au coeur de notre quotidien, il est aussi au coeur des inégalités, parce que c'est le logement qui plombe le pouvoir d'achat. Les dépenses de logement ne cessent d'augmenter, et davantage pour les plus pauvres, avec 30 % à 40 % de charges mensuelles. La question du logement est donc au coeur des inégalités et votre politique interroge. Une politique du logement, c'est d'abord du sens, porter des convictions et, en premier lieu, celle de la réduction des écarts. Pour moi, elle doit s'appuyer sur deux piliers : la mixité et la diversité ; la mixité sociale et la diversité des produits au sein d'un même territoire.

Le logement d'abord, tout le monde peut être d'accord, monsieur le ministre, mais attention, en même temps, aux questions sociales, spatiales, de plus en plus nombreuses. Je m'interroge sur votre politique de la ville : les quartiers ne peuvent être coincés entre accès au logement et paupérisation. Quelle mixité, quelle solidarité, sachant que les quartiers ont été les plus impactés par la pandémie, comme vous l'avez dit dans ce combat contre les inégalités par le logement, aggravées par la pandémie, quelles sont vos propositions pour la mixité sociale et quelles mesures envisagez-vous de prendre ? La parole est à M. le ministre. Je profite

comme vous le savez, concernent la rénovation thermique des bâtiments. Il s'agit d'une thématique essentielle, puisqu'elle permet d'associer économie, emploi, justice sociale, objectifs climatiques et réduction de la dépendance énergétique de notre pays. Il est important de rappeler dans cet hémicycle que pour plus d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que nous entrons dans une crise économique et sociale majeure, la rénovation thermique est aussi une question de lutte contre les inégalités, après que la crise sanitaire a amené des millions de millions de ménages à se confiner dans un habitat indigne. Face à ces enjeux, la Convention citoyenne pour le climat propose notamment une interdiction de location des passoires énergétiques étiquetées F et G à partir de 2028. Cette proposition est assortie d'une obligation de rénovation globale permettant d'atteindre une performance serait sanctionné par un malus sur la taxe foncière et elle s'accompagnerait d'un renforcement et d'une simplification des aides à la rénovation, notamment pour les propriétaires modestes.

à un renforcement des moyens alloués à la rénovation énergétique, afin d'allier relance et écologie. Si cette ambition budgétaire est louable, il faut non seulement qu'elle soit à la hauteur de l'enjeu mais aussi qu'elle s'accompagne de mesures contraignantes : la seule incitation n'a jusqu'à présent pas suffi. Alors que se multiplient les appels à construire un « monde d'après » juste et solidaire, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, comment votre ministère accueille ces propositions fortes, issues des citoyens, et quelle place il souhaite leur donner dans les débats à venir ? La parole

fortes et ambitieuses, à la fois exigeantes quant aux objectifs climatiques et soucieuses de justice sociale. C'est bien le type de mesures dont nous avons besoin pour affronter l'urgence environnementale à laquelle nous sommes confrontés, mais aussi pour

Face à cette crise, le Gouvernement a réagi, en mettant en place un dispositif de chômage partiel, en accordant des aides exceptionnelles aux entreprises et aux autoentrepreneurs, en versant une aide exceptionnelle de solidarité, mais aussi, ce qui a un lien direct avec notre débat, en allongeant de plus de trois mois, jusqu'au 10 juillet prochain, la trêve hivernale. Cependant, l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense depuis le début d'avril une forte hausse des appels vers la ligne dédiée

de retour à la normale ne présage pas des évolutions à venir, qui dépendront de la conjoncture, il témoigne en tout cas de l'effet qu'ont eu les mesures du Gouvernement pour amortir les effets de la crise. Pour poursuivre ces efforts, des acteurs tels que la Fondation Abbé Pierre demandent des mesures, en particulier un moratoire des loyers, et des moyens supplémentaires sous la forme d'un fonds national d'urgence d'aide à la quittance

Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat font de la rénovation énergétique des logements un sujet de premier plan. Les logements que l'on appelle communément des « passoires énergétiques » constituent un problème qui n'est pas seulement écologique. effet, la rénovation énergétique efficace de nos bâtiments a aussi des bénéfices en termes sociaux, économiques et sanitaires. C'est un levier de relance inéluctable pour nos entreprises, notre artisanat et nos territoires, mais aussi un levier pour le pouvoir d'achat des Français et pour la création d'emplois ainsi qu'une impulsion nouvelle pour l'Europe, qui voit dans la rénovation énergétique un sujet majeur. Beaucoup d'engagements ont été pris depuis le Grenelle de l'environnement, mais nous avons aujourd'hui besoin d'une vraie accélération dans ce domaine pour combler notre retard. Pour cela il nous faut simplifier et compléter nos dispositifs pour les rendre plus lisibles et plus efficaces. Cela nous permettra d'avoir une approche tant performante que rapide. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions en la matière ? Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser la place que prendraient les bailleurs sociaux dans un tel dispositif ?

Aussi, le plan de relance doit passer en priorité par la construction et la rénovation énergétique efficace des bâtiments, vecteur important d'activité économique.

Monsieur le ministre, combien ce dispositif a-t-il coûté aux finances publiques pour un résultat aux trois quarts inefficace ? Il faut faire évoluer les procédures et les contrôles pour que ces moyens financiers écologiques soient correctement utilisés. Pour que les Français rénovent et investissent, il faut de la confiance. Ils doivent s'assurer que l'investissement dégagera un gain financier à moyen ou long terme. Les plateformes de rénovation énergétique et les conseillers des espaces info énergie sont des outils fiables. Il faut que l'État soutienne plus fortement et plus durablement ces dispositifs

de la construction, auquel le secteur du logement est intimement lié, représente plus de 6 % de l'emploi et subit de plein fouet les conséquences de la crise que nous traversons. Il représente également 20 % des émissions de gaz à effet de serre. À travers ces deux chiffres, il est facile de comprendre les perspectives offertes par ce secteur, qu'il convient de soutenir pour relancer l'économie tout en y inscrivant des solutions environnementales fortes. Je souhaite aussi rappeler que différents textes législatifs ont défini le logement décent et ont introduit des exigences d'isolation thermique et de performance énergétique. L'Ademe estime d'ailleurs que les travaux d'isolation permettraient de réaliser jusqu'à 25 % d'économie sur la facture énergétique annuelle des ménages. Je crois que nous pouvons tous convenir que la rénovation des logements est partie prenante de tout plan de transition écologique. Il faut aussi s'assurer,, que que les exigences existantes seront appliquées. S'agissant des surfaces, rappelons qu'un logement en location est défini comme devant disposer, au moins, d'une pièce principale de 9 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 2,20 ce type de logement ressemble plus à un dortoir qu'à un logement digne de la France du XXI siècle ! D'ailleurs, la crise sanitaire a aussi révélé l'importance que revêtent les critères de qualité d'un logement souvent transformé en bureau par le télétravail. Je plaide donc pour une incitation forte à la réhabilitation et à la rénovation énergétique des bâtiments, mais j'ai aussi la conviction que nous devons nous atteler à la « reconception » du parc immobilier, dès lors que des travaux sont engagés, car la rénovation doit non pas se résumer à son volet énergétique, mais être plus globale. Dans ce contexte, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il faille, d'une part, redéfinir ce qu'est un logement décent, en France, en 2020, et, d'autre part, accompagner les propriétaires et instaurer, peut-être, une obligation de rénovation énergétique du logement, comme celle qui existe déjà pour les bâtiments tertiaires ?

dépend directement des bailleurs sociaux, qui sont des acteurs majeurs de la construction et de la rénovation de logements. Or, en touchant le secteur du bâtiment, la crise a provoqué un retard de trois mois dans leurs travaux : aujourd'hui, seuls 69 % des chantiers affichent un niveau d'activité pleine. Les bailleurs sociaux sont pourtant des moteurs de la relance économique, en vertu de leur relation avec les territoires. Bien avant la crise, leur situation financière avait été fragilisée par les décisions du Gouvernement prises depuis deux ans. Pour rappel, la réduction de loyer de solidarité (RSL), décidée à la suite de la baisse des APL, a fortement affecté leurs ressources et les a obligés à puiser dans leurs fonds propres.

C'est tout un écosystème qui attend que l'État redevienne un acteur du financement du logement social et le garant de la solidarité nationale. Il est donc plus que nécessaire de revenir sur les réformes qui ont mis les bailleurs sociaux en difficulté : reconnaître le logement social comme un bien d'utilité publique avec une TVA à 5,5 à 5,5 %, revaloriser les APL, bloquer la RLS à son niveau actuel et, par conséquent, abandonner le palier d'augmentation prévu pour 2022. Monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous apporter à ces légitimes demandes ? La parole est à M. le ministre.

en abondant le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) en lieu et place d'Action Logement- il ne peut pas se décharger sur d'autres organismes de ses responsabilités -et les fonds de solidarité pour le logement. L'État doit également être un garant de la solidarité nationale en sécurisant l'accès des particuliers au logement, en rétablissant l'APL accession et le prêt à taux zéro

le devenir de 80 % de notre territoire, même s'il ne représente plus que 20 % de la population. Je souhaite aborder le bâti rural et le logement dans ces mêmes territoires, qui sont en permanence oubliés, quand ils ne sont pas tout simplement condamnés par la loi.

au quotidien. Dans le même temps, la loi doit permettre de développer l'urbanisme dans les territoires ruraux en supprimant un certain nombre de règles et en adaptant le code de l'urbanisme. Certes,

le ministre, allons-nous enfin donner une chance à ces territoires en adaptant le code de l'urbanisme, en y protégeant mieux les activités agricoles, nécessaires à l'entretien de l'espace rural pour construire et réhabiliter le bâti existant ?

qui se dressent sur le chemin menant aux multiples objectifs environnementaux, tous plus ambitieux les uns que les autres, que nous inscrivons régulièrement dans le marbre des textes législatifs. Nous nous accordons aussi globalement sur l'urgence de la situation. Par conséquent, de toutes les démarches utiles, il me semble que nous devrions privilégier les plus efficientes.

Dans le cadre du groupe de travail « Enseignement supérieur » que j'ai piloté au nom de la commission de la culture, mes collègues et moi-même avons recommandé un plan de rénovation des bâtiments universitaires, facteur à la fois de relance économique sur le plan local et de démarche écologique, en écho aux propos qu'a tenus le Président de la République le 14 juin dernier. Avec ses 18,6 millions de mètres carrés, dont un tiers est classé passoire énergétique, le parc immobilier universitaire est un gros consommateur d'énergie. Les simulations d'ores et déjà effectuées à partir d'un échantillon d'universités expérimentales démontrent que la rénovation des campus induit une réduction de charges très importante. Là où la rénovation globale des logements est encore difficile à mettre en place, celle des bâtiments publics peut et doit être un levier d'action. Les universités sont prêtes à s'engager dans de tels investissements, qui permettent de créer des emplois, de soutenir le secteur du BTP et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. votre gouvernement est-il prêt à élaborer des contrats de plan État-université pour la rénovation des bâtiments universitaires ? est à M. le ministre. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir m'excuser de n'avoir pas pris connaissance de votre document, ce que je ferai avec grand plaisir : je n'ai donc pas en tête le détail des propositions que vous formulez et je ne voudrais pas m'engager par

assez loin des incantations idéologiques qu'on a pu entendre récemment et qui ont peut-être pour vocation unique de braquer les acteurs et,, de maintenir le.

puisque le secteur du bâtiment représente 43 % de la consommation d'énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre. Il répond ensuite à un enjeu social, puisque 12 millions de nos concitoyens sont en situation de précarité énergétique. Le médiateur national de l'énergie a d'ailleurs signalé une hausse significative des interventions pour impayés de factures d'énergie en 2019. Il répond enfin à un enjeu économique. On recense ainsi en France 7,5 millions de passoires énergétiques : autant de chantiers non délocalisables en perspective pour lancer fortement ce secteur fondamental dans notre économie, celui du bâtiment et des travaux publics. Le Président de la République a annoncé le 14 juin dernier un plan de modernisation du pays, notamment autour de la rénovation thermique des bâtiments. Cette ambition nécessite une implication forte de l'État à une tout autre échelle que les politiques menées ces dernières années. Nous savons tous que le de la rénovation n'a pas eu lieu : on peut même dire que la France piétine sur ce chantier pourtant majeur. Aussi les parlementaires socialistes proposent-ils d'engager une approche nouvelle de la rénovation thermique des bâtiments en créant immédiatement une prime unique pour le climat. Cette prime universelle aurait pour objectif d'accompagner l'ensemble des propriétaires du parc privé dans la réalisation de travaux améliorant significativement la performance énergétique du logement. Elle permettrait de préfinancer jusqu'à 100 % des coûts de rénovation thermique en fonction des ressources des ménages.

le reste à charge, qui est souvent trop élevé. Troisième frein, la multiplicité des aides à la rénovation. C'est pourquoi la prime pour le climat prévoit aussi de fusionner les différents dispositifs existants afin de les rendre plus lisibles et accessibles. Monsieur le ministre, nous vous proposons ce dispositif, construit avec les apports des principaux acteurs du logement au travers de nombreuses auditions, pour un véritable changement d'échelle de la rénovation énergétique dans notre pays. Vous en saisirez-vous pour accompagner concrètement le plan de modernisation annoncé par le Président de la République ? La parole est à M. le ministre.

Si j'étais taquin, je dirais qu'entendre le groupe socialiste prôner la prime et non pas le crédit d'impôt

M. Philippe Pemezec. Monsieur le ministre, devenir propriétaire de son logement est un excellent moyen de se prémunir contre les aléas de la vie. Cela permet aussi de se constituer un patrimoine et, si on le souhaite, de laisser un héritage à ses enfants.

Malheureusement, monsieur le ministre, la loi ÉLAN est une véritable usine à gaz ! Tout d'abord, il aura fallu attendre plus d'un an les décrets d'application.

Au lieu de simplifier le système, on l'a complexifié ; je pense en particulier à la publicité et à la procédure de vente des logements sociaux. pour se porter acquéreur, il faut être le plus rapide et le premier à répondre à une annonce publiée sur une plateforme internet, sans examen préalable des dossiers ni analyse des situations ou de leur degré d'urgence

perte d'activité, perte de productivité, surcoûts importants et persistants, bouleversement des chantiers, décalage des plannings, survie. Le BTP est en effet l'un des secteurs qui a vu son activité se réduire mois d'avril dernier, soit le même taux que l'hôtellerie-restauration, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative. La reprise est là, mais progressive et fragile. Des chantiers du bâtiment ont redémarré au cours du mois de mai dernier. Néanmoins, l'activité des entreprises n'a pas encore retrouvé son rythme normal normal : une entreprise sur trois n'a pas retrouvé un niveau d'activité habituel. Certes, votre gouvernement a pris des mesures de soutien en faveur du bâtiment, telles que les prêts garantis par l'État, l'activité partielle et un fonds de solidarité, pas moins que nos entreprises du bâtiment attendent des actes suffisants dans le soutien à l'investissement local et dans la réactivité, dans un contexte où l'instruction des permis de construire s'est arrêtée. Aussi, les exonérations de charges prévues dans le PLFR 3 doivent être étendues pour que nombre d'entreprises n'ayant pas subi de chute d'activité supérieure à 50 % au cours de la période allant du 1 février au 31 mai soient éligibles. Si ce n'est pas le cas, cette mesure sera d'effet très limité. L'accroissement de la dotation de soutien à l'investissement local est insuffisant : le milliard d'euros fléchés sur l'investissement local dans la transition écologique ne compensera pas les 9 milliards d'euros de baisse de recettes fiscales locales, attendues avant la fin de l'année. En outre, les mesures d'incitation à l'investissement local Enfin, une valorisation du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est primordiale, afin d'inciter à l'investissement local. Monsieur le ministre, les entreprises du bâtiment et de l'artisanat ont besoin de confiance dans leur relance. Quelles mesures supplémentaires proposez-vous pour susciter cette confiance ?

La situation du secteur de l'immobilier, chacun l'a dit ici, est d'une gravité extrême. Les chiffres dont nous disposons, monsieur le ministre, proviennent du secteur privé, non de votre ministère.

Rappelons-nous que, trois mois après le déclenchement de la crise des, un plan de relance de la primo-accession à la propriété dans le neuf avait été engagé sous l'impulsion

Cette fois-ci, quatre mois après le début de la crise, on commence seulement à se préoccuper d'un plan pour le bâtiment ! J'espère que l'administration des finances-

notamment en accélérant les délais et les conversions de bureaux en logements. Vous avez dit à plusieurs reprises, monsieur le ministre, que, si rien ne repart, c'est parce que les banques ne font pas preuve de bonne volonté. C'est un peu facile

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le bilan de l'application des lois

chargé des relations avec le Parlement, qui répondra au nom du Gouvernement aux questions du Sénat. Cela fait maintenant près d'un demi-siècle que le Sénat fait du contrôle de l'application des lois votées une priorité dans son contrôle de l'action du Gouvernement. Chaque année, le Sénat affine le périmètre de son contrôle. Les commissions suivent attentivement la parution des décrets d'application et celle des rapports au Parlement, mais d'autres problématiques entrent désormais dans le champ de notre contrôle. Nous vous avions notamment interpellé l'année dernière, monsieur le ministre, au sujet des ordonnances. La crise sanitaire que nous avons traversée a remis cette question au coeur de l'actualité. Nous avons voté dans les mois passés des dizaines d'habilitations, dont toutes n'étaient peut-être pas dictées par des nécessités d'urgence ou d'ordre technique rendant difficile un examen selon la procédure législative normale. Très récemment, la suppression de nombreuses habilitations du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et leur inscription directe dans notre droit en vigueur l'ont d'ailleurs illustré. Le Parlement peut légiférer rapidement et efficacement. Cette tentation de la facilité est donc difficilement acceptable. La présidente Valérie Létard l'avait relevé l'an dernier : les délais dans lesquels interviennent les ordonnances sont généralement supérieurs au délai moyen d'adoption d'une loi. L'argument de la célérité n'est pas toujours confirmé par les faits, et nous pouvons également le vérifier en comparant les délais imposés au Parlement pour l'examen de certaines lois et ceux dans lesquels interviennent leurs mesures d'application.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Le bilan de l'application des lois constitue un temps fort du contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement. Il permet de s'assurer que les textes d'application sont pris en temps et en heure et qu'ils respectent la volonté du législateur. Les commissions permanentes sont au fondement de ce dispositif. Tout au long de l'année, elles mènent un travail approfondi de veille réglementaire pour les textes d'application relevant de leur compétence. Ce suivi a dû cette année être effectué dans des conditions délicates du fait de la crise sanitaire. Je remercie donc vivement les commissions, qui se sont mobilisées pour continuer à assurer le suivi de l'application des lois.

Cette réforme accentue le rôle des commissions, en confiant au rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi la responsabilité du suivi de son application. Il est encore trop tôt pour tirer les conséquences de cette évolution, qui doit permettre d'améliorer le contrôle de la publication des mesures réglementaires. L'efficacité du bilan de l'application des lois découle également d'un dialogue nourri avec les différentes administrations, ainsi qu'avec le secrétariat général du Gouvernement. Cet échange a fait la preuve de son efficacité, comme en témoigne l'accroissement notable du nombre de décrets publiés quelques jours à peine après les différentes communications des commissions sur le sujet. Le bilan que je vous présente aujourd'hui analyse la mise en application des lois adoptées lors de la session parlementaire 2018-2019, c'est-à-dire entre le 1 octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Durant cette période, 49 lois ont été votées, dont 22 étaient d'application directe. Fait notable, la proportion de lois résultant d'une initiative parlementaire est particulièrement élevée cette année : près de la moitié des lois de la session sont ainsi issues de propositions de loi. Le taux global d'application des lois est de 72 %, soit un taux légèrement inférieur à celui de la session précédente, où il était de 78 %. Sur les 918 mesures réglementaires attendues, seules 660 ont été publiées. Je regrette d'autant plus ce recul que, si la prise des mesures d'application a été perturbée par la crise sanitaire, elle ne concerne en réalité que peu les textes prévus par les lois adoptées au cours de la dernière session. En effet, le Gouvernement s'engage depuis 2008 à prendre les décrets d'application six mois au plus tard après la parution des lois. Ce délai était déjà écoulé au début de la crise sanitaire. Il y a un an, je me félicitais de la réduction du délai nécessaire à la prise des mesures d'application. Ce constat ne peut malheureusement être réitéré cette année. En moyenne, les textes réglementaires ont été publiés cinq mois et douze jours après la promulgation de la loi, soit près d'un mois de plus qu'au cours de la précédente session. Les raisons de ce retard sont parfois liées à des difficultés juridiques apparues notamment lors des consultations obligatoires, de la notification à la Commission européenne, ou éventuellement du passage en Conseil d'État. L'objectif de ce bilan annuel est précisément de permettre au Gouvernement d'expliciter les raisons qui conduisent à l'absence de mise en application de certaines lois. Cependant, le recours à la procédure accélérée est toujours généralisé et concernait 31 lois sur la session 2018-2019. Par conséquent, il est essentiel que la mise en application complète des lois soit à la hauteur de la rapidité exigée du législateur. Les principaux points de vigilance demeurent ceux qui avaient été soulevés en 2019. Le rendu des rapports est notamment chroniquement insuffisant : comme les années précédentes, le taux de dépôt de dépôt des rapports sur la session est très bas. Il se situe à 12 % à peine, contre 35 % l'année passée. Il n'est de plus que de 27 % sur la législature. La faiblesse du taux de remise des rapports est encore moins compréhensible s'agissant des rapports demandés par le Gouvernement lui-même : seuls 8 % des rapports prévus par un amendement gouvernemental ont été remis depuis 2017. À croire que ce type de disposition avait pour seule vocation avait pour seule vocation de donner une satisfaction de principe à une demande, sans réelle volonté d'aboutir. Le Sénat a de son côté effectué d'importants efforts pour limiter les demandes de rapports aux seuls cas où ceux-ci sont indispensables à l'information du Parlement. Mes collègues reviendront sans doute sur ce point pour les rapports relevant de la compétence de leur commission. Les raisons pour lesquelles certains décrets ne sont pas publiés sont parfois confuses. À titre d'exemple, alors que ce sujet avait déjà été évoqué il y a un an, deux textes essentiels pour la gouvernance d'Action Logement et figurant dans la loi portant

partenaires réunissant élus et opérateurs du logement social, prévu par un décret de mai 2019, n'est pas paru. Pouvez-vous nous expliciter les raisons de l'absence de publication de ces deux textes, qui limitent grandement la réforme de la gouvernance de cet organisme ? Pour ma part, compte tenu de l'allongement du délai nécessaire à leur parution, j'ai peine à croire que celui-ci soit dû à de simples raisons techniques. Cet exemple illustre également les différences d'interprétation dans nos méthodes de décompte des textes d'application.

J'en viens maintenant à la question des ordonnances, que nous avions déjà largement évoquée lors du précédent bilan. Le sujet est plus que jamais d'actualité, pour deux raisons de nature différente. Tout d'abord, plus d'une cinquantaine d'ordonnances ont été prises pendant la crise sanitaire. Il y a un an, vous nous aviez indiqué, monsieur le ministre, qu'au cours des six dernières années le nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance était supérieur au nombre de lois adoptées par le Parlement. Pour autant, je réitère le constat effectué lors de ce débat l'argument de rapidité avancé pour justifier l'utilisation d'ordonnances ne tient pas. En effet, le délai moyen entre la promulgation de la loi d'habilitation et la publication des ordonnances est de près d'un an, soit un délai supérieur au temps moyen d'adoption de la loi. De nombreuses habilitations sont encore non utilisées. Je n'en citerai qu'un exemple : l'article 17 de la loi pour un État au service d'une société de confiance habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures pour renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Cette ordonnance devait être publiée avant avril 2019, mais le Gouvernement a depuis indiqué y avoir renoncé. Par ailleurs, la ratification des ordonnances n'est pas toujours effective, faute d'inscription des projets de loi de ratification à l'ordre du jour des assemblées. Depuis de longues années, cela prive le Parlement d'un débat sur la conformité de l'ordonnance à la volonté du législateur. La décision du Conseil constitutionnel du 28 mai dernier, dite « Force 5 », a donné une nouvelle dimension à cette préoccupation sur la portée du débat parlementaire, en indiquant qu'une ordonnance non ratifiée acquiert une valeur législative à compter de la fin du délai d'habilitation dès lors qu'elle intervient dans le domaine de la loi.

Les conséquences de cette décision sont doubles. Il est plus nécessaire que jamais pour le Parlement de veiller en amont à la définition précise du périmètre de l'habilitation consentie au Gouvernement. Et quelle sera désormais la portée exacte de la ratification parlementaire ? Si nous souhaitons éviter que le Parlement ne perde la main sur l'élaboration de la loi, il me semble que l'examen des lois de ratification doit être pleinement intégré dans un agenda parlementaire déjà extrêmement dense. À l'heure actuelle, les projets de loi de ratification une fois déposés ne sont que rarement examinés, faute d'inscription à l'ordre du jour. Monsieur le ministre, comment comptez-vous organiser l'inscription à l'ordre du jour des projets de loi de ratification, indispensables à la poursuite du débat parlementaire et au plein exercice de la fonction de contrôle ? En application de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Toutefois, si le dépôt du projet de loi de ratification est quasi systématique, rien ne contraint le Gouvernement à inscrire son projet à l'ordre du jour des assemblées. Un réexamen de cette règle ne s'impose-t-il pas ? Le Gouvernement compte-t-il désormais indiquer dès la demande d'habilitation à à quelle date il entend inscrire le projet de loi de ratification à l'ordre du jour ? Prévoit-il ce véritable échéancier, comme c'est le cas pour les mesures d'application des textes adoptés ? Cela éviterait de courir un risque supplémentaire de se voir refuser une demande de légiférer par ordonnances. J'ai souhaité mettre l'accent cette année sur le suivi de l'application des expérimentations, qui sont de plus en plus fréquemment utilisées dans la construction de la loi. Plus d'une centaine d'expérimentations ont été mises en oeuvre au cours de ces deux dernières années. Elles peuvent être de formidables outils, en garantissant plus de souplesse et une meilleure adaptation aux circonstances locales, à condition que leur suivi soit effectif. Je regrette toutefois des défauts récurrents dans le suivi et la généralisation des expérimentations. Ainsi, plus du quart d'entre elles est abandonné en cours de mise en oeuvre. De même, des généralisations précoces d'expérimentation, parfois sans même attendre les premières évaluations, sont encore trop nombreuses. C'est par exemple le cas de l'expérimentation sur le relèvement du seuil de revente à perte prévue par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales

je voudrais tout d'abord remercier Mme Valérie Létard, l'ensemble des présidents de commission, ainsi que les services du Sénat de leur travail toujours minutieux, sur la base duquel nous allons échanger cet après-midi. Alors que, l'an passé, le rapport soulignait que le taux d'application résultant des calculs du Sénat était « proche de celui du Gouvernement », cette année, ce sont plutôt nos divergences méthodologiques qui sont mises en exergue, avec des taux qui, en première analyse, peuvent paraître très divergents : 82 % pour le Gouvernement, contre 72 % pour le Sénat. Nous avons de longue date une méthodologie différente ; vous l'avez d'ailleurs souligné, madame la sénatrice. Premièrement, le Gouvernement ne retient que les mesures immédiatement applicables, le Sénat y ajoute les mesures différées, ce qui conduit à un différentiel d'environ 150 mesures. Deuxièmement, le taux que nous vous présentons ne prend pas en compte les arrêtés. Le Premier ministre est le titulaire du pouvoir réglementaire. Il est donc naturel qu'il assure un suivi général de l'application des lois et que nous venions en débattre chaque année avec vous. Cela permet d'avoir une vision « panoramique » des quelque 1 600 décrets qui sortent chaque année. Par comparaison, le nombre d'arrêtés réglementaires pris chaque année est d'environ 8 000. Par définition, les arrêtés sont signés par chaque ministre compétent, mais rarement par le Premier ministre. Outre la difficulté qu'il y aurait pour le secrétariat général du Gouvernement (SGG) à suivre entre deux et quatre dizaines d'arrêtés chaque jour, il s'agit là de la responsabilité de chaque ministre. Un ministre est par nature responsable pour suivre en continu les arrêtés qu'il doit prendre. La modification du règlement du Sénat du 6 juin 2019, qui confie au rapporteur d'un texte le suivi de son application, doit de notre point de vue permettre le suivi fin de ces arrêtés.

Il convient toutefois de souligner que le nombre de mesures à prendre a significativement augmenté, d'environ 55 % ! Nous sommes passés de 461 mesures pour 2017-2018

pour être honnête intellectuellement, on constate un recours plus systématique sous cette législature et la précédente que sous la XIII législature. Cela n'est sans doute pas sans lien avec la révision de la Constitution de 2008, qui a profondément modifié les règles de fixation de l'ordre du jour : à défaut de procédure accélérée, un texte déposé depuis moins de six semaines ne peut être inscrit à l'ordre du jour, ce qui, à un ou deux jours près, peut conduire à retarder son examen d'un bon mois. Les conditions d'examen exceptionnelles que nous avons connues au cours des trois derniers mois ne sont pas représentatives, je le crois, de la manière dont l'examen des textes s'est déroulé depuis 2017. Et même si le Gouvernement demande généralement

c'est dire ce qu'étaient la situation au début des années 2000 et le chemin qui a été parcouru par l'ensemble des gouvernements depuis lors ! La situation a désormais radicalement changé ; entre 80 % et 90 % des mesures sont prises dans un délai de six mois. Dans les faits, le Parlement sera prochainement destinataire, dans le délai de six mois, de 100 % des tableaux faisant le point sur cette application. Nombre d'administrations peuvent ainsi avoir le sentiment que les tableaux qu'elles remplissent et qui sont transmis au Parlement répondent à l'objet de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004. La transmission de ces tableaux vaut-elle transmission du « rapport » au sens de cet article ? C'est en effet la question que pose l'évolution de la situation.

Il est parfois tentant de bouleverser ce séquençage. J'ai souvenir des débats que nous avions encore récemment lors de l'examen de la loi portant diverses dispositions urgentes au sujet de l'expérimentation de relèvement du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions. La solution qui a été retenue par la commission mixte paritaire et définitivement adoptée par le Parlement me paraît de ce point de vue conforme à l'objectif d'approfondissement des évaluations que vous appelez de vos voeux. Vous m'interrogez en outre sur les ordonnances. Leur nombre varie de

pour reprendre le mot de Jean-Marc Sauvé lors d'un colloque de 2014 sur la législation déléguée, me semble difficile à contester. Je ne crois pas qu'il faille y voir une forme de facilité à laquelle céderaient les gouvernements, quels qu'ils soient, et

empirique l'analyse de l'ancien vice-président du Conseil d'État : « L'inflation législative [ ...] a trouvé dans la législation déléguée un exutoire durable, d'abord, pour répondre à l'urgence de certaines réformes ou pour décharger le Parlement de l'adoption de textes techniques [ ...], ensuite, pour investir très largement le domaine devenu très extensif de la loi Vous avez évoqué la décision que le Conseil constitutionnel a rendue consacrant le caractère législatif d'une ordonnance non ratifiée après l'expiration du délai d'habilitation.

combien le calendrier parlementaire est contraint et ne peut accueillir l'examen d'une quarantaine de projets de loi supplémentaires chaque année, sauf à considérer cette ratification comme une simple formalité. cette ratification comme une simple formalité. Enfin, le Gouvernement envisage une évolution de la gouvernance d'Action logement, pour faire suite à une série de dysfonctionnements. Dans ce cadre, il a demandé un rapport à l'inspection générale des finances, afin de vérifier que les règles de gouvernance sont respectées, de faire des recommandations pour les améliorer, de détailler les implications que l'absence de mise en oeuvre de ces règles peut avoir. L'adoption de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la gouvernance du groupe a donc été suspendue. Dans l'intervalle, des réunions informelles entre les élus et les opérateurs du logement social peuvent naturellement être organisées, dans l'attente d'une refonte globale du cadre réglementaire.

sur l'application des lois, la fameuse loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dite « loi OTSS », tant attendue par les professionnels de santé, n'était applicable qu'à hauteur de 30 %. Aucune des onze ordonnances prévues dans le texte, sur des sujets aussi lourds d'enjeux que les autorisations sanitaires ou l'organisation des hôpitaux de proximité, n'avait été publiée.

de solliciter du Parlement des habilitations à légiférer par ordonnance sur des projets de réforme à l'état d'ébauche, qui n'ont été ni muris ni concertés ni élaborés plus avant.

Pour autant, un certain nombre de textes seront publiés avec retard. La loi du 23 mars 2020 a d'ailleurs reporté de quatre mois le terme de toutes les habitations en cours prévues par la loi OTSS. Le récent projet de loi portant diverses dispositions urgentes prévoit également le report de la réforme du deuxième cycle des études médicales, ainsi que d'autres habilitations : certifications périodiques des médecins, emploi médical hospitalier. Le Ségur de la santé doit tirer les conséquences de la crise sanitaire. Vous avez d'ailleurs vous-même posé la question des réglementations à adopter. Il faudra transformer les métiers, revaloriser ceux qui soignent, définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins, simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes et fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Hormis les textes à caractère technique, le Ségur de la santé va nécessairement impliquer que les projets de textes à prendre en application de la loi OTSS soient revus à cette aune. C'est d'ailleurs un peu ce à quoi vous nous invitez. Il en

l'énergie et au climat, ou loi Énergie-climat, connaît un début d'application extrêmement difficile, avec, à la date du bilan établi par la commission, une dizaine de mesures réglementaires publiées sur environ 70 décrets ou arrêtés prévus, une ordonnance prise sur cinq articles et 15 habilitations, aucun rapport formellement remis au Parlement sur les six attendus du Gouvernement. Un quart des ordonnances aurait déjà dû être publié, la ministre de la transition écologique et solidaire ayant indiqué devant notre commission faire usage de la prolongation de quatre mois des délais permise par la loi d'urgence sanitaire. ministre, il y a pire que le retard. Pour ce qui concerne la programmation pluriannuelle de l'énergie, certains objectifs sur le biogaz, l'hydrogène ou l'éolien en mer ne sont pas ceux adoptés par le législateur. Cela constitue un dévoiement inacceptable de l'esprit de la loi. Ce constat est regrettable compte tenu des objectifs énergétiques et climatiques ambitieux visés dans cette loi,

d'Action logement. Derrière cette question technique, c'est la pérennité de la mission et du groupe paritaire qui est en jeu. Notre pays fait face à une crise économique majeure. Il faut donner les moyens à Action logement de fonctionner normalement. J'ai bien compris qu'une inspection était en cours, mais c'est

la crise sanitaire explique une partie de ces retards dans la publication des mesures d'application. La majorité des textes à prendre dans le délai de six mois sont des décrets en Conseil d'État, avec une phase de consultation obligatoire au cours des mois de février et mars, notamment en Commission de régulation de l'énergie ou encore le Conseil supérieur de l'énergie, et la saisine du Conseil d'État au cours des mois de mars et avril, pour une publication au plus tard au mois de mai 2020. La période de confinement de deux mois a donc conduit à décaler le calendrier. Toutefois, je peux d'ores et déjà vous indiquer que le décret relatif à l'autorité environnementale a été examiné par la section des travaux publics du Conseil d'État le 16 juin 2020 et devrait être publié prochainement que le décret relatif aux aides pour l'électrification rurale est en cours de transmission au Conseil d'État. Les travaux se poursuivent par ailleurs. Les textes concernant les garanties d'origine du biogaz représentant six mesures d'application sont en cours de consultation, avec une perspective de saisine du Conseil d'État en juillet. Les mesures sur la fin des tarifs réglementés de vente de gaz et les fournisseurs de dernier recours, qui concernent sept mesures, ont été mis dans le circuit des consultations. Sur les 16 ordonnances prévues par cette loi, 4 ont été prises, les autres ont vu le terme de leur habitation prorogé de quatre de quatre mois par la loi du 23 mars dernier. Six habilitations feront l'objet d'ordonnances qui devraient être examinées en conseil des ministres au mois de juillet prochain. Elles portent sur l'adaptation du droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat, sur les procédures du comité de règlement des différends

l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la gouvernance du groupe a été effectivement suspendue. Il est vrai que le délai est long et que la volonté du Gouvernement est désormais d'aller assez vite. Je ne peux pas vous donner une date, mais je relayerai vos préoccupations auprès de Julien Denormandie.

adopté dix-neuf conventions internationales, et nous avons poursuivi la mise en application des lois des sessions antérieures. Bien entendu, ce que nous suivons avec le plus d'attention, c'est la mise en oeuvre

92 %, ce qui, deux ans après, peut être considéré comme satisfaisant. Il manque deux arrêtés, mais qui sont d'importance mineure. Le Gouvernement pourrait améliorer ces statistiques, puisque nous restons bloqués à 83 % d'application. Mais il y a toujours ce fameux décret de la loi de juillet 2010 sur l'allocation au conjoint d'un agent au service étranger qui manque à l'appel ; j'imagine que ce sont plus des questions juridiques et financières qui bloquent ce dispositif. Nous le rappelons chaque année. année. Autre élément de satisfaction, on constate un net progrès dans la transmission des rapports, notamment pour tout ce qui relève des opérations extérieures et intérieures. Pour la première fois, cela a été transmis. Nous vous en remercions. La parole est à M. le ministre.

conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent civil de l'État en service à l'étranger qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire ». Ce dispositif avait pour vocation de remplacer l'actuel supplément familial versé directement à l'agent expatrié lorsque son conjoint se trouve dans une situation similaire à celle qui est prévue dans le texte de 2010. La mise en oeuvre de cette nouvelle allocation s'est toutefois heurtée à deux principales difficultés ; vous en avez d'ailleurs évoqué au moins une. sur le plan technique, il n'est pas possible d'indemniser sur le titre II une personne pour laquelle il n'existe aucun lien juridique avec l'État. D'autre part, la direction générale des finances publiques et la direction de la sécurité sociale ont une interprétation différente- c'est le sujet juridique que nous avons devant nous -du régime social appliqué à cette nouvelle allocation.

pendant la crise sanitaire, le poids important de la commande publique militaire dans notre tissu industriel et la nécessité de nous préparer correctement aux crises de tous ordres que nous voyons émerger dans le monde et qui pourraient encore survenir sont autant d'éléments qui nous conduisent à rester fidèles à nos engagements pris collectivement pour nos armées en 2018.

Au 31 mars 2020, le taux d'application était acceptable, de l'ordre de 60 %. Nous avons eu l'occasion d'échanger par écrit sur le calendrier des contenus des mesures restant à prendre avec le Secrétaire général du Gouvernement, ainsi qu'avec Jean-Michel Blanquer. pas. Sur les quatre autres textes, je constate que la mise en oeuvre des deux lois d'initiative parlementaire se révèle particulièrement difficile. La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information n'a à ce jour démontré ni son efficacité ni sa pertinence. Le Sénat s'était d'ailleurs fermement opposé à son adoption, tout comme à celle plus récemment, de l'article 1 de la loi Avia contre la haine en ligne, justement censuré jeudi dernier par le Conseil constitutionnel. La loi relative à la rémunération des journalistes et éditeurs sur les plateformes en ligne au titre des droits voisins se trouve, quant à elle, privée de son applicabilité par le refus des plateformes de se conformer à la loi. On ne peut que le déplorer. Ces textes montrent les limites de l'action législative nationale face au secteur de l'internet. Pour en sortir, nous suggérons de s'appuyer enfin sur les travaux sénatoriaux et les propositions de résolution européenne pour

Je souhaiterais néanmoins savoir à quelle date le rapport annuel faisant état du montant des fonds recueillis pour cette reconstruction, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation sera transmis au Parlement. Quel est le calendrier retenu pour la parution des ordonnances permettant de déroger au droit commun dans le cadre des travaux de restauration ? Le délai d'habilitation prévue par la loi expire en effet le 29 juillet 2020.

De plus, l'article 8 de cette même loi prévoit que l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale publie chaque année un rapport ayant le même objet. Ce rapport sera publié avant la fin de l'année 2020. d'habilitation des ordonnances que vous avez évoquées a été prolongé de quatre mois par la loi du 23 mars, ce qui porte la date du terme de l'habilitation au 29 novembre 2020. Un projet d'ordonnance a été examiné lors d'une réunion interministérielle le 10 mars dernier. L'opportunité de déroger aux dispositions applicables dans certains domaines, aux travaux de restauration de la cathédrale et d'aménagement de son environnement immédiat est toujours en discussion, afin de bien identifier les dispositions effectivement applicables au chantier auxquelles les dérogations seront réellement nécessaires. Une deuxième réunion interministérielle en date du 15 juin a permis d'envisager le calendrier suivant : la rédaction du texte pour début juillet 2020, la concertation avec la mairie de Paris courant juillet, la saisine du Conseil d'État fin août 2020, enfin la présentation en conseil des ministres à la mi-octobre de la même année. Le premier décret d'application manquant de la loi relative à la création de l'Agence nationale du sport, qui est relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport, a été transmis au Conseil d'État le 22 juin 2020. Le second, qui concerne le délégué territorial de l'Agence nationale du sport, devrait également être transmis au Conseil d'État au cours de cette semaine. Une publication de ces deux textes pourrait ainsi intervenir avant la fin du mois de juillet 2020.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mes questions portent sur l'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Nous avions consenti à examiner ce texte dans l'urgence et à maintenir des habilitations à légiférer par ordonnance sur des sujets majeurs, à condition que les choix retenus par le Gouvernement soient ensuite discutés. Or aucune des quatre ordonnances prises sur le fondement de cette loi n'a été ratifiée par le Parlement, et l'examen des projets de loi de ratification n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée.

n'a pas été tenu. Par ailleurs, un certain nombre de réserves importantes ont été formulées par le régulateur sur cette ordonnance. À cela s'ajoutent des incertitudes, puisque le cadre juridique de l'ouverture à la concurrence n'est toujours pas finalisé. Ce manque de visibilité pour les nouveaux entrants, les salariés et les régions est de nature à nuire à l'ouverture à la concurrence. Et le Gouvernement n'a toujours pas pris l'ordonnance visant à tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accord collectif. À la suite de l'échec des négociations relatives à l'accord sur les classifications et les rémunérations en février dernier, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari nous avait indiqué que l'État tiendrait parole et prendrait l'ordonnance prévue.

Pourquoi ce délai ? Quand ce décret sera-t-il publié ? Enfin, qu'en est-il de la publication du décret relatif aux modalités de transfert de certaines petites lignes aux régions ? Même si ce transfert est prévu par la loi d'orientation des mobilités, et non par le nouveau pacte ferroviaire, il est essentiel dans le cadre de l'ouverture à la concurrence.

des décrets manquants de cette loi, le premier porte sur la composition et les moyens de fonctionnement d'une instance commune. Il était subordonné à la signature d'un accord relatif aux conditions d'exercice social entre les entreprises issues du groupe public ferroviaire, ce qui a été fait par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives à la fin de l'année 2019. Le projet de décret a été finalisé et doit maintenant être examiné décret concerne la portabilité de la garantie d'affiliation au régime général de retraite de la SNCF en cas de changement d'employeur. Le projet de décret reste en attente des orientations en matière de réforme globale des retraites.

À la suite de l'échec de la négociation collective sur les classifications et rémunérations, le Gouvernement a décidé qu'il pourrait utiliser cette ordonnance afin d'établir un cadre commun en la matière pour les salariés de la branche ferroviaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la session écoulée, la commission des finances constate un taux d'application des lois en progrès, mais elle regrette l'allongement des délais de publication. Moins du tiers des textes réglementaires ont été publiés dans les six mois. La raison de ce retard réside notamment dans les délais de réponse aux demandes introduites auprès de la Commission européenne en matière d'aides d'État. Pas moins de sept mesures d'application de la loi de finances initiale pour 2019 sont ainsi en attente. Monsieur le ministre, le Gouvernement pourrait-il à l'avenir présenter dans son rapport d'application des lois un état des lieux précis des demandes introduites auprès de la Commission européenne concernant des aides d'État ? le président de la commission des finances avait largement évoqué l'an passé les retards dans l'application de la loi relative à la lutte contre la fraude. Les textes réglementaires sont désormais pris, mais nous en surveillerons très précisément la mise en oeuvre concrète. Il reste cependant les articles 14 et 15, qui octroient aux agents des douanes et de l'administration des impôts un droit de communication des données de connexion pour les enquêtes portant sur les délits douaniers et fiscaux les plus graves. Une question préjudicielle posée par l'Estonie est pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne. Compte tenu de l'importance d'accorder des moyens supplémentaires à la lutte contre la fraude, pouvez-vous nous confirmer que les décrets sont prêts à être publiés dès que la décision de la Cour sera connue, c'est-à-dire à l'été, nous dit-on ? Et nous y sommes ! Autre sujet plus ponctuel : l'article 134 de la loi de finances pour 2012 relatif au régime de licence de vente du tabac dans les départements d'outre-mer. L'entrée en vigueur de cette disposition a été repoussée au gré des lois de finances jusqu'au 30 juin 2019, sans pour autant que la mesure entre en application. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ne faut-il pas reconnaître que ce dispositif n'est pas applicable ? Comptez-vous au contraire le mettre en oeuvre rapidement ? Enfin, le Sénat a adopté le 21 avril dernier un taux réduit de TVA pour les tenues de protection, sujet cher à notre rapporteur général. Lors de son audition devant la commission des finances, le 11 juin, le ministre Bruno Le Maire répondait en ces termes : « Le taux réduit de TVA, qui a été voulu par le Président de la République, doit être mis en oeuvre rapidement. Un arrêté est en cours de signature. » Pourquoi cet arrêté n'est-il toujours pas pris ? La parole

relative à la lutte contre la fraude, les projets de textes ont été retirés de l'examen du Conseil d'État le 28 mars 2019 à la suite d'une question préjudicielle estonienne en cours d'instruction à la Cour de justice de l'Union européenne. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 15 octobre 2019.

S'agissant de l'application de l'article 134 de la loi de finances pour 2012, je rappelle que la mise en place d'un dispositif d'encadrement de la vente au détail du tabac manufacturé dans les départements et régions d'outre-mer par l'attribution de licences de vente a été plusieurs fois reportée. L'avis très défavorable émis par les assemblées délibérantes de ces collectivités, qui estiment ne pas pouvoir mettre en oeuvre cette réforme, en est la principale raison. Cette opposition s'explique par la difficulté à disposer des moyens humains et financiers nécessaires à l'attribution des licences et par la crainte d'une forte incidence sur le tissu économique, notamment pour les petits commerces, qui occupent outre-mer une place importante dans le réseau de distribution du tabac manufacturé. Si l'objectif de santé publique est indiscutable, ces réserves nécessitent de poursuivre une réflexion partagée avec les collectivités concernées sur les moyens engagés pour lutter contre le tabagisme. Ces territoires ne doivent naturellement pas figurer en retrait de la lutte contre le tabagisme. À ce stade, la réflexion s'oriente vers un assouplissement

et de réforme pour la justice, qui fait suite d'ailleurs à une disposition législative de 2016 sur la République numérique, qui concerne l'open data des décisions de justice. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous retrouver dans le labyrinthe administratif pour saisir ceux qui devraient prendre ce décret le plus rapidement possible ? Nous en avons besoin constatons enfin une tendance de plus en plus forte à recourir aux ordonnances. La décision récente du Conseil constitutionnel nous inquiète. Monsieur le ministre, allez-vous continuer à inscrire à l'ordre du jour prioritaire les projets de loi ratifiant les ordonnances,

enregistrons un taux d'application des lois moins satisfaisant que les années précédentes. Au 31 mars 2020, le Gouvernement a comptabilisé 106 mesures prises sur les 156 à prendre, soit un taux d'application de 68 %. Au 23 juin, ce taux s'élève à 82 %, puisque 25 nouvelles mesures ont été appliquées depuis le 31 mars. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique appelle 94 mesures actives, dont 77 sont appliquées à ce jour, ce qui porte le taux d'application de la loi à 82 %. Ce taux était de 57 % au

le 7 mai dernier. S'agissant du décret d'application de l'article 49, le Conseil d'État a été saisi du projet de décret en février, après que celui-ci a été validé lors d'une réunion interministérielle à la fin du mois de décembre 2019 et que toutes les consultations obligatoires ont été réalisées en janvier. L'examen en section, initialement programmé le 24 mars, a dû être reporté en raison des mesures de confinement. Il s'est tenu en avril. Dans le cadre d'une visioconférence, le décret a ensuite été publié le 6 mai. Enfin, pour ce qui concerne le décret relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives du 19 mars 2020, il a été décidé de suspendre sa publication, qui n'apparaissait pas opportune dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, compte tenu de l'ampleur des conséquences sur le fonctionnement des juridictions. Cette suspension de publication a été dernièrement levée, de telle sorte que le projet de décret qui est en cours de contreseing devrait être publié d'ici à la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les résolutions européennes dont la commission des affaires européennes est à l'initiative sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution donnent au Gouvernement des orientations pour les négociations avec les vingt-six autres États membres et les institutions européennes. Le rapport que j'ai présenté au mois de février dernier démontre la réelle influence de la Haute Assemblée à Bruxelles. En effet, dans 87 % des cas, nos résolutions européennes ont été prises en compte au cours des négociations. Elles influent donc directement sur le contenu des directives et des règlements finalement adoptés, et par conséquent sur la législation française. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en matière européenne passe également par un dialogue étroit et fructueux avec la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, avec qui notre commission débat de façon interactive sur le suivi de nos résolutions, et avec le secrétariat général aux affaires européennes, qui nous fournit des informations très complètes, même si je les souhaiterais plus régulières tout au long de l'année. Au-delà du contrôle sur les négociations que mène le Gouvernement à Bruxelles, la mission de la commission des affaires européennes a été étendue l'an dernier. Précisément, la commission s'est vue confier à titre expérimental en février 2018 une mission d'alerte

En mai dernier, le secrétaire général du Gouvernement m'avait assuré de l'engagement de l'exécutif à lutter de manière générale contre les surtranspositions, ajoutant qu'il était à notre « disposition pour tenter de trouver un moyen de mieux remédier aux surtranspositions dans les ordonnances, qui est un point important de l'action normative du Gouvernement ». Je voudrais donc connaître l'état de la réflexion du Gouvernement pour progresser dans cette voie. Un calendrier a-t-il d'ores et déjà été arrêté pour définir une méthode de travail associant la commission des affaires européennes ? La parole est

entreprises et les citoyens. C'est d'ailleurs bien sur ce sujet que vous nous alertez, monsieur le président. Afin de lutter contre ces surtranspositions, le Premier ministre a publié dès le 26 juillet 2017 une circulaire qui proscrit par principe toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive, sauf à ce qu'elle fasse l'objet d'un choix assumé et confirmé par le Premier ministre. Le principe de cette circulaire est applicable dans le cadre de la préparation des décrets, des projets de loi et des projets d'ordonnance. Parallèlement à ces règles visant à prévenir de nouvelles surtranspositions, la circulaire précitée entendait réduire le stock en s'appuyant sur un travail d'inventaire confié à une mission d'inspection. Sur la base de cet inventaire, le Gouvernement a initialement présenté un projet de loi portant

initialement contenu dans les articles 19 à 22 du projet de loi. Enfin, pour les mesures qui n'ont pu être reprises à ce stade dans un projet de loi thématique, la suppression de la surtransposition interviendra dès qu'un vecteur législatif approprié sera disponible, notamment dans le cadre de futurs travaux de transposition qui permettront de supprimer d'anciennes surtranspositions.

l'école occupe une place singulière au sein des institutions de notre pays. Elle conditionne la promesse républicaine. Notre histoire nous l'enseigne ; le présent nous le rappelle. Si la réforme de l'école figurait déjà au coeur de l'action du Gouvernement, elle apparaît désormais aussi comme l'un des points névralgiques de la gestion de la crise inédite que traverse notre pays. C'est pourquoi je souhaite vous interroger au sujet de l'application de la loi pour une école de la confiance en général, et de ses dispositions relatives à l'inclusion des enfants handicapés, en particulier.

En second lieu, pouvez-vous nous garantir que les diverses dispositions réglementaires qui concernent les élèves en situation de handicap et ceux qui souffrent de trouble du langage ou de difficultés psychologiques seront prises d'ici à la rentrée 2020- nous espérons que celle-ci se déroule dans de meilleures conditions ? Je pense notamment aux articles 13, 30 et 31 de ladite loi, qui traitent respectivement du dépistage des troubles du langage et des apprentissages chez les enfants de moins de six ans, de la coopération entre établissements médicosociaux et scolaires pour la prise en charge des élèves en situation de handicap et de l'accompagnement des jeunes qui présentent des difficultés psychologiques. La parole est à M. le ministre.

un groupe de travail composé de toutes les parties prenantes a été constitué. Ses travaux, interrompus par la crise sanitaire, vont reprendre dans les prochains jours avec l'objectif de produire le projet de décret en octobre. Deux consultations sont à prévoir : celle, obligatoire, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et celle, facultative, mais au fond incontournable, du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Concernant le décret d'application de l'article 31 de la loi relatif au fonctionnement en dispositif intégré des établissements scolaires et médicosociaux pour les jeunes en situation de handicap, un groupe de travail a également été constitué. Il va reprendre ses travaux, avec un

et, sous réserve du délai de nouvelle convocation en cas de vote unanime défavorable, soumis ensuite au contreseing. de vote unanime défavorable, soumis ensuite au contreseing. Enfin, pour ce qui est de l'arrêté prévu à l'article 46 de la loi relatif au cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap, le groupe de travail créé poursuit ses travaux. Une quatrième réunion est prévue ce jeudi 25 juin pour valider le cahier des charges. Trente heures de formation seraient notamment dédiées à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Un arrêté sera ensuite publié en septembre 2020, de telle sorte que les prochaines formations répondront bien au cahier des charges.

du texte de ratification, l'ordonnance ne peut être modifiée que par la loi. Le Conseil se borne donc à constater que, dès ce moment, elle a acquis une valeur législative. C'est la Constitution

assemblées s'étaient émues de ne pas voir inscrites à l'ordre du jour des ratifications d'ordonnances. Je me permets d'appeler l'attention du président Bas un instant,

assez varié des propositions de loi déposées par les deux assemblées, aucune ne revient jamais sur le contenu des ordonnances, alors que les opportunités seraient multiples. On peut aussi procéder par voie d'amendement. Le président Bas et moi-même l'avons fait tout récemment

l'usage des caméras mobiles par les sapeurs-pompiers et les surveillants pénitentiaires. Utilisées depuis 2013 par les forces de police et de gendarmerie, les caméras mobiles ont pour finalité de sécuriser les interventions de ces agents publics confrontés dans l'exercice de leurs missions à une agressivité croissante. Les événements récents témoignent, si besoin en est, de la pertinence de ce dispositif. La loi du 3 août 2018 pérennise également l'utilisation des caméras mobiles par les agents des polices municipales. La loi renvoyait la définition des modalités d'utilisation des caméras mobiles et des enregistrements visuels collectés à trois décrets en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Tous ces décrets ont été pris au-delà des six mois. Le premier, pour les agents de police municipale, a été publié le 27 février 2019. Le deuxième, pour les sapeurs-pompiers, a, quant à lui, été pris le 17 juillet 2019. La publication du troisième, pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, date du 23 décembre 2019. Il aura donc fallu attendre seize mois après la promulgation de la loi pour que puisse commencer une expérimentation amenée à durer trois ans, alors que nous partageons tous tous l'intérêt d'un tel dispositif. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que l'amélioration de la rapidité de l'application des lois constitue l'un des moyens pour restaurer la confiance et l'intérêt des Français pour la chose publique ? En ce

Tous les professionnels nous le disent, la présence de la caméra incite certaines personnes à davantage maîtriser leurs actes et leurs propos ; elle renforce donc la sécurité de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers et de nos surveillants pénitentiaires. Les enregistrements effectués facilitent l'identification et la poursuite des auteurs d'agressions verbales ou physiques ; ce sont des preuves utiles pour la justice. Depuis 2013, cet équipement utilisé par les forces de l'ordre a su démontrer son efficacité.

notre initiative, un rapport sur la relance des trains de nuit dans le cadre de la discussion de la loi d'orientation des mobilités et alors que ce rapport doit être remis avant le 30 juin, quand pourrons-nous, monsieur le ministre, en disposer ? Comment les parlementaires seront-ils associés à la mise en oeuvre de la relance du ferroviaire, alors que les enjeux écologiques sont encore plus prégnants

à cette loi que « l'État étudie le développement de nouvelles lignes [ ...], en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d'une amélioration de l'offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés

Conformément aux orientations de cette loi, le ministère de la transition écologique et solidaire étudie jusqu'au 30 juin le développement des nouvelles lignes de trains d'équilibre des territoires. Cette étude concerne aussi bien le jour que la nuit. Concernant la nuit, la première phase de l'étude a consisté à réaliser une comparaison avec les autres réseaux européens qui sont dans une logique de redéveloppement des trains de nuit- Autriche, Suède, Norvège. Un échange approfondi a notamment eu lieu avec les chemins de fer autrichiens qui sont à la pointe dans ce domaine. Des échanges se sont également déroulés avec différents constructeurs, le matériel roulant constituant un élément clé pour l'exploitation de telles lignes. Quatre segments de marché ont été identifiés pour établir des liaisons de nuit potentielles : relations intérieures ou internationales entre grandes agglomérations, relations entre chapelets de villes, dessertes touristiques saisonnières et dessertes d'aménagement du territoire. Le rapport de cette étude technique devrait être disponible dans les prochains jours.

centraux sur ces questions, ainsi que des associations. Ces auditions sont nécessaires pour valider les résultats de l'étude technique. Il est proposé de les organiser au début de l'automne selon des modalités à définir et de transmettre par la suite l'ensemble de ces éléments au Parlement.

le taux d'application des lois est dans l'ensemble satisfaisant, bien qu'en léger retrait par rapport à la session précédente. Cependant, il est décevant pour certains textes pourtant jugés clés par le Gouvernement, tels que la loi relative à l'organisation et à la transformation du système transformation du système de santé ou les articles relatifs à la privatisation d'ADP contenus dans la loi dite Pacte. Depuis le début de la crise du Covid-19, le Parlement s'est attelé à adopter des textes prioritaires dans les plus brefs délais. Il est temps que l'État en fasse de même, afin d'apporter de la visibilité aux différents acteurs, parfois mis à rude épreuve- je pense notamment à la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cela pose encore une fois la question du rôle du Parlement, ce qui m'amène aux deux principaux sujets de ma question. d'abord, l'accroissement du recours aux ordonnances soulève un véritable problème démocratique, surtout lorsqu'aucune urgence ne le justifie, car le délai entre la demande d'habilitation et la prise de l'ordonnance est supérieur au délai moyen de vote d'une loi. Ensuite, le taux de remise des rapports demandés par le Parlement au Gouvernement est très faible. Pis encore, il a chuté par rapport à la session précédente : alors qu'il était de 35 % l'an passé, il atteint désormais 12 %.

Monsieur le ministre, pour redonner au Parlement sa place dans le débat, pouvez-vous nous préciser la ligne du Gouvernement concernant le recours aux ordonnances et le retard pris quant à la remise des rapports demandés ? La parole Monsieur le ministre,

de rapports remis en application de la loi du 9 décembre 2004. Ces rapports remis dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi mentionnent les textes réglementaires et les circulaires publiés pour la mise en oeuvre de ladite loi.

et des tableaux de suivi. Même si le Sénat estime que cela ne suffit pas à satisfaire entièrement l'obligation de la loi de 2004, c'est une avancée qui permettra, me semble-t-il, d'assurer un meilleur suivi. Encore une fois, je crois que le travail bilatéral entre les rapporteurs et les ministères pourra fournir des compléments qualitatifs utiles à ces tableaux de suivi.

rédiger un texte de loi est gratifiant et, disons-le, réserver certains points techniques, parfois hasardeux, au pouvoir réglementaire peut être confortable. Face à ce constat, nous avons chacun une part de responsabilité. Néanmoins, la difficulté de l'État à prendre en temps et en heure les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois contraste avec des délais toujours plus courts plus courts imposés au Parlement. La procédure accélérée semble être devenue la norme et les ordonnances se multiplient. En faisant ce constat, comme beaucoup, je m'interroge. Sous couvert d'un environnement économique et juridique toujours plus pointu,

Rien n'est pire pour nuire à la confiance dans l'action publique qu'un texte sans portée. Rien n'est pire pour la démocratie que lorsqu'elle ressemble à un bavardage. D'ailleurs, ne dit-on pas que, lorsque la loi bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite ? Ce bilan n'est pas technico-juridique ; c'est celui du fonctionnement de notre démocratie. Sachons le regarder tel qu'il est et souvenons-nous de ces milliers de gilets jaunes qui ne croyaient plus en rien ! La parole est à M. le ministre.

je constate que le monde est devenu d'une incroyable complexité, et notre droit n'en est finalement que le reflet. Gardons-nous de penser que la simplification du droit est la solution à tout, même s'il doit rester intelligible. Nous pouvons sans doute faire plus simple, mais nous risquons alors

évidemment pas d'accord avec vous. L'application de la loi peut faire l'objet d'un contrôle par le juge administratif, lequel peut même engager la responsabilité de l'État pour absence de prise d'actes réglementaires d'application d'une loi. De plus, le Gouvernement est pleinement responsable devant le Parlement ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis avec vous, cette année encore, pour débattre de l'application des lois.